et assurément républicaines. Ne l'oublions pas, le but même d'une association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, pour reprendre les mots de 1789. En miroir, le but de toute association est de faire vivre le lien et la passion de ceux qui ont décidé de se retrouver pour avancer ensemble. Là où la solidarité peut parfois s'effacer, l'association prend la place ; là où la force publique faillit, l'association prend le relais.

le 12 mai dernier, la commission des lois a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Cet examen a été conduit selon la procédure de législation en commission, prévue aux articles 47 à 47 du règlement du Sénat. Sénat. Vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, ce texte a une histoire assez longue puisqu'il a été déposé par vous-même et certains de vos collègues députés sur le bureau de l'Assemblée nationale, en octobre 2018 ; le Sénat l'a adopté en première lecture en en juillet 2019. C'est un long parcours, mais il ne faut jamais baisser les bras ; la preuve : nous sommes là aujourd'hui. Ainsi que je l'ai indiqué en commission, le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture répond au souhait que le Sénat avait exprimé de préserver

Si nous avons dû proposer des modifications, le 12 mai dernier, c'est pour des raisons de pure cohérence législative et, je pense pouvoir le dire, ce texte fait aujourd'hui l'objet d'un consensus.

le Sénat avait refusé d'inscrire dans la loi la possibilité, pour les associations, de conserver un « excédent raisonnable » correspondant à tout ou partie d'une subvention non utilisée. C'est là-dessus que nous avons travaillé et que nous avons trouvé un point d'équilibre. Dans la même logique, le Sénat avait supprimé l'article 1 , qui prévoyait une obligation de versement des subventions accordées

L'Assemblée nationale a ainsi maintenu la suppression de l'article 4 empêchant les communes de faire usage du droit de préemption sur les biens cédés à titre gratuit aux associations ayant la capacité de recevoir des libéralités.

tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée ». Cette rédaction, issue d'une coconstruction, donnera, je pense, satisfaction à tout le monde. L'article 1 a également fait l'objet d'une nouvelle rédaction, afin de prévoir que le délai de versement d'une subvention à une association

Tout en maintenant le souhait de permettre aux associations de bénéficier de facilités de trésorerie et d'une plus grande prévisibilité sur le versement des subventions qui leur ont été allouées, ces nouvelles rédactions préservent les compétences des collectivités. Elles reposent sur la compréhension des difficultés que peuvent avoir les associations. Nous avons trouvé le bon

que ce projet de loi donne satisfaction à un amendement adopté par le Sénat en première lecture sur l'alignement des obligations de transparence financières pour toutes les associations qui gèrent une activité cultuelle, il impose le contrat d'engagement républicain- un objectif que nous partagions -aux associations sollicitant des subventions publiques. C'est une réforme que nous avons approuvée et qui permettra de lutter contre certaines dérives que l'on a pu constater dans une partie

c'est au terme d'une procédure législative particulièrement longue que nous allons enfin pouvoir apporter une réponse aux plus de 1,3 million d'associations que compte notre pays ; ces structures attendent d'être soutenus, après la crise sanitaire qui a mis en berne la vie associative dans notre pays. C'est tout l'intérêt de cette proposition de loi, enrichie tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qui doit faciliter le fonctionnement et le développement des associations d'un point de vue financier. Cette nécessité se fait de plus en plus pressante à l'heure de la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire

de la sortie de crise sanitaire, que les associations doivent être soutenues. Ces dernières sont des actrices essentielles de la vie des Français et leurs efforts ne doivent pas avoir été faits en vain. À cet égard, je tiens à saluer Mme la rapporteure pour la qualité de son travail depuis le début du parcours de cette proposition de loi. En outre, la qualité de la relation entre notre rapporteure et son homologue de l'Assemblée nationale a permis de protéger les intérêts que nous défendons au Sénat, démontrant la volonté de nos deux chambres d'aboutir à un texte ambitieux, au service des associations mais également des collectivités. À ce titre, le groupe Union Centriste se réjouit que la plupart des dispositions introduites par la Haute Assemblée

En tant que partenaires privilégiées de la vie sociale, les communes ne doivent pas se voir imposer des contraintes disproportionnées, voire contreproductives, ayant pour conséquence d'alourdir inutilement leur travail de coopération avec les associations.

Le groupe Union Centriste partage les dispositions introduites au cours de la navette et considère que cette proposition de loi va dans le bon sens, pour plusieurs raisons. Premièrement, ce texte multiplie les sources de financement des associations, en autorisant les prêts entre associations d'un même réseau. Deuxièmement, il simplifie les relations entre les autorités administratives et les associations ; nous savons à quel point les démarches administratives sont un frein à l'efficacité et à la rapidité des mesures. D'une part, une autorisation sera accordée aux associations de conserver une partie d'une subvention non dépensée ; d'autre part, le texte ouvrira aux fondations la possibilité d'être agréées pour enseigner la conduite.

des comptes de campagne n'ayant pas été attribués dans le délai prévu. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce texte. La parole

aura finalement animé les débats. Plusieurs dispositions ont déjà fait l'objet d'une adoption conforme- les prêts entre associations, l'identification des comptes inactifs -, donc il est temps de conclure. C'est le souhait partagé par l'ensemble du Mouvement associatif et c'est la raison pour laquelle notre groupe n'a pas déposé d'amendements sur ce texte. La crise sanitaire

En 2020, selon le Mouvement associatif, 30 000 associations sont menacées de disparition, 55 000 ont déclaré ne pas pouvoir maintenir les salaires et l'on décompte 60 000 emplois en moins. Les déclarations d'embauche ont chuté de 45 % et les créations d'association de 40 %. les adhésions ont décru de 25 % à 50 % dans les associations sportives, culturelles et de loisirs. C'est l'hécatombe, douloureux reflet des difficultés qui sont devant nous. Les 16 millions de bénévoles et de salariés que comptent nos associations sont- vous l'avez vous-même rappelé, madame la secrétaire d'État -une richesse exceptionnelle pour notre démocratie. Cette proposition de loi qui vise à faciliter le fonctionnement et le développement de ces associations sur le plan financier doit désormais être adoptée. Toutefois, l'esprit de consensus que j'évoquais ne constitue pas un blanc-seing donné au Gouvernement ; cette proposition de loi doit être vue pour ce qu'elle est : un petit pas visant à prendre en compte les attentes d'un secteur associatif en difficulté. En reprenant des demandes du secteur ainsi que des mesures adoptées sous le précédent quinquennat, notamment notamment dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté, chère au coeur de Patrick Kanner, mais censurées par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi va dans le bon sens. L'examen de ce texte intervient dans un contexte de crise, mais également de désengagement complet de l'État par rapport au milieu associatif. La suppression de plus de 250 000 contrats aidés en deux ans, la réduction de la dotation globale de fonctionnement et, plus largement, la baisse générale de la collecte grand public ont entamé le processus de délitement du secteur associatif, privant les associations de leur capacité d'embauche et certaines personnes d'une réinsertion sociale par le biais de l'emploi.

aux jeunes, notamment aux enfants et aux adolescents. Nous espérions une grande loi pour le secteur associatif, mais nous n'oublions pas que celui-ci a grandement besoin de ces premières mesures, qui sont urgentes. Donc, ne ralentissons pas leur adoption.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe Les Indépendants - République et Territoires. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes tous attachés au monde associatif : les associations jouent un rôle essentiel et irremplaçable. Dans nos villes, nos quartiers et nos villages, au plus près des habitants de toutes les générations, elles sont utiles au quotidien. C'est encore plus vrai aujourd'hui, dans la période difficile que nous traversons bien sûr, aux associations du secteur sanitaire et social, mais également à celles qui facilitent la continuité pédagogique ou qui aident à lutter contre le décrochage scolaire. Dans cette situation inédite, les associations ont prouvé leur pertinence. Nous pouvons donc être fiers du dynamisme de notre secteur associatif. On estime à 1,5 million le nombre d'associations en France. Dans le département dont je suis élu, le Nord, où l'on en compte près de 48 000, l'engagement citoyen est très actif. Le monde associatif, c'est aussi plus de 70 000 créations par an, 16 millions de bénévoles et 1,8 million d'emplois, à temps plein ou partiel. C'est enfin un budget total de 113 milliards d'euros, soit l'équivalent de 3 % du produit intérieur brut (PIB). Ces derniers chiffres sont éloquents pour exprimer la place que les associations occupent dans la vie économique de notre pays. Néanmoins, leur rôle essentiel ne se résume pas à cet aspect, il va bien au-delà. Je veux parler ici des valeurs qu'elles portent : celles de l'engagement, des solidarités, de la philanthropie et de la générosité. Aussi, soutenir les associations paraît indispensable, car elles sont au coeur de la cohésion sociale. La proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, soumise à notre vote aujourd'hui, est en navette depuis plus de deux ans. Elle est issue d'une proposition de loi que vous aviez déposée en octobre 2018, madame la secrétaire d'État, lorsque vous étiez députée. composé initialement de six articles, a été réécrit et étoffé par nos deux chambres. Je me félicite que le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ait tenu compte des enrichissements apportés par le Sénat afin de préserver l'équilibre entre associations et collectivités territoriales. Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 1 définissant désormais les conditions dans lesquelles une association peut conserver « tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée dans le cadre d'une convention signée entre une collectivité et une association. Je me réjouis qu'elle ait abandonné la notion trop imprécise d'« excédent raisonnable La rédaction de l'article 1 a également été modifiée afin que le délai de versement d'une subvention à une association soit « fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l'autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n'ait arrêté d'autres dates de versement ou n'ait subordonné le versement à la survenance d'un évènement déterminé Enfin, je suis satisfait du maintien de la suppression de l'article 4 privant les communes d'utiliser le droit de préemption urbain sur les biens immobiliers cédés à titre gratuit aux associations et fondations. En effet, ce droit, très encadré, est nécessaire à la cohérence des projets d'urbanisme des collectivités. Avant de conclure, je tiens à rendre hommage, à cette tribune, aux millions de femmes et d'hommes, bénévoles associatifs, qui agissent avec l'élan du coeur et ne comptent pas leur temps. Madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, mes chers collègues, les associations font vivre le tissu économique local et dynamisent la vie de nos communes rurales et de nos quartiers urbains. Simplifier leur gestion et alléger la tâche de ceux qui s'y consacrent est un objectif que le groupe Les Indépendants partage pleinement. Il votera donc bien évidemment en faveur de cette proposition de loi.

loi a eu le rare honneur de ne pas subir une procédure accélérée et de croiser d'autres textes structurants, comme la loi de finances pour 2020 créant un Fonds pour le développement de la vie associative, le fameux FDVA. issu d'une large concertation entre les secteurs divers du monde associatif, tels que le sport, l'environnement, le social, la culture, et les acteurs institutionnels impliqués, a abouti à 59 propositions concrètes. La France compte environ 1,3 million d'associations au sein desquelles sont engagés 16 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Un point auquel je suis tout particulièrement attaché, ainsi que mon groupe, est la place primordiale des associations dans le monde de l'économie sociale et solidaire Oui, la forme associative est celle qui est le plus souvent choisie- près de 90 %, d'après l'de 2015 -pour encadrer l'exercice d'une activité qui s'inscrit dans le cadre ambitieux des solidarités. Je ne rappellerai pas combien les écologistes encouragent et soutiennent un engagement citoyen fort, sur l'ensemble des territoires et dans l'ensemble des domaines. Nul besoin, non plus, de rappeler qu'avec la crise du covid-19 les associations ont encore plus montré qu'elles étaient précieuses pour les plus précaires, les plus isolés, les plus démunis et les plus abandonnés. La sécurisation du financement des associations, en particulier dans leurs relations avec les collectivités territoriales, constitue le cadre le plus structurant pour assurer la pérennité de ces acteurs du quotidien. ce gouvernement n'aura pas épargné les associations par sa politique fondée sur la théorie des premiers de cordée, dite aussi du ruissellement, par la baisse des subventions publiques, la fin des contrats aidés, sans oublier le tout récent contrat d'engagement républicain. Comment, alors, s'étonner des baisses de création et d'adhésion aux associations ? Pour en revenir à l'étude des articles qui restaient en discussion après ce long processus législatif, nous avons pu nous pencher sur l'équilibre nécessaire entre, d'une part, les contraintes financières qui s'imposent aux associations, et, d'autre part, leurs contraintes administratives, tout particulièrement dans leurs relations avec les collectivités territoriales. L'article 1, qui reprenait la proposition 50 du rapport de 2018, a abandonné la notion « d'excédent raisonnable », pour définir les fonds issus de subventions publiques qu'une association pourra conserver d'une année sur l'autre. Si j'entends que cette notion est trop vague, le fait d'indiquer qu'une association pourra conserver « tout ou partie » de ces fonds dans le cadre de conventions signées avec une collectivité s'éloigne des recommandations initiales du rapport. Ainsi, dans le cadre de ces conventions, cela laisse la place au dialogue pour définir les conditions dans lesquelles l'association peut conserver « tout ou partie » de ces montants. Il convient tout de même de poser la question des différences territorialisées de ces conditions de trésorerie, voire des différences qui pourraient être faites d'une association à l'autre. À ce titre, j'ai déjà alerté cette assemblée de l'importance de permettre aux petites structures associatives de l'ESS, dont l'activité dépend parfois d'une tarification publique ou de subventions pour des délégations d'action, de mettre en réserve une partie de leur résultat d'exploitation. La souplesse et la visibilité de leur gestion sont au coeur de la pérennité de ces structures. Cette mesure serait tout à fait bienvenue pour les petites associations issues de l'ESS. Nous saluons l'adoption d'un délai légal de versement des subventions de soixante jours, qui permet aussi une plus grande visibilité à la vie associative. Les modifications apportées par les articles 3 A et 3 B sur la dévolution des excédents des comptes de campagne électorale se révèlent un signal fort : sans action du mandataire ou de l'association de financement électoral sur le devenir de l'excédent, ce dernier reviendra au FDVA. C'est la reconnaissance du rôle essentiel des associations dans la vie locale. L'article 3 intègre d'ailleurs les parlementaires dans le collège consultatif du FDVA. Je salue la position de notre commission sur l'article 5, qui a adopté la modification portée par le groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ayant souhaité inscrire le rapport prévu dans cet article dans une temporalité plus longue. Cela permettra vraisemblablement d'avoir une réelle analyse de l'impact de la suppression de l'impôt de Dans l'ensemble, ce texte, comme celui étudié en parallèle par la commission de la culture, va dans le bon sens, celui d'une reconnaissance des associations, de leur travail et d'une simplification de leur fonctionnement, y compris au niveau de leur trésorerie. conscient de l'importance de la place des associations dans notre société dans tous les domaines de la vie quotidienne, et malgré quelques réserves, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera ce texte. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe

Ce texte que vous portiez, madame la secrétaire d'État, comme auteure puis rapporteure lorsque vous siégiez à l'Assemblée nationale, est le fruit d'un long travail de concertation mené en lien avec le Mouvement associatif. Il reprend notamment plusieurs dispositions qui n'avaient pas pu être intégrées, en 2017, dans le périmètre de la loi Égalité et citoyenneté. L'entrée en vigueur de ce texte, qui répond à la nécessité de permettre aux associations d'affermir leur stabilité par le recours à de nouvelles ressources, est donc très attendue par le monde associatif. C'est justement pour répondre à cette impatience et parce que nous savions que certaines de ses dispositions étaient très attendues que, avec le groupe RDPI l'initiative d'Alain Richard, nous avons fait le choix de reprendre, au sein de la loi améliorant la justice de proximité et de la réponse pénale, la possibilité pour l'État de mettre à disposition des associations, fondations ou organismes d'aide au logement des biens immobiliers saisis lors de procédures pénales. Grâce à cette initiative, ce dispositif est effectif depuis le mois dernier. La deuxième lecture n'a donné lieu en commission des lois qu'à de simples ajustements de portée rédactionnelle ou de coordination, et n'a pas altéré sur le fond le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Et pour cause, l'Assemblée nationale s'est elle-même montrée bienveillante envers les réserves que le Sénat avait pu exprimer en première lecture et les a intégrées dans son travail. Elle a ainsi répondu à la nécessité de préciser la définition de l'« excédent raisonnable

tels que l'élargissement de la liste des associations pouvant bénéficier de l'excédent du compte de campagne ou le maintien de la possibilité, pour les communes, de faire usage du droit de préemption sur des biens cédés à titre gratuit aux associations. Ainsi, le texte que nous nous apprêtons à voter préserve utilement l'équilibre des liens établis entre collectivités territoriales et associations. Comme les collectivités, les associations ont oeuvré au soutien des populations les plus fragiles durant la crise sanitaire. Si le secteur associatif a été au coeur de la crise sanitaire, il a lui-même été gravement éprouvé par son contexte. Les chiffres sont saisissants :-40 % de création d'association et-25 % d'adhésions dans les associations culturelles et sportives. Aussi, ce texte initialement conçu pour soutenir un secteur en pleine mutation est aujourd'hui rendu nécessaire pour soutenir son redémarrage et promouvoir le retour vers l'engagement. Concrètement, la proposition de loi permettra aux associations de bénéficier de facilités de trésorerie et d'une plus grande prévisibilité sur le versement des subventions, grâce à la possibilité pour l'association de conserver tout ou partie de la subvention qui n'aurait pas été intégralement dépensée. Elle permettra également aux associations de s'accorder mutuellement des prêts de trésorerie, sans intérêt, pour une durée inférieure à deux ans. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une politique à plusieurs niveaux. Je pense ainsi aux moyens engagés pour soutenir le secteur dans le cadre du plan France Relance et, notamment, au plan exceptionnel de soutien de 100 millions d'euros pour les associations de prévention et de lutte contre la pauvreté. Complétant utilement ces dispositifs, le présent texte a fait l'objet d'un large consensus sur nos travées, à l'issue d'un travail constructif dont nous espérons qu'il aboutira prochainement. Dans cette perspective, le groupe RDPI votera la proposition de loi.

là où l'État, parfois, ne le fait plus. Nous devons d'autant plus nous pencher sur leur sort que nombre d'entre elles n'ont pas été épargnées par la crise et ont vu leur activité ralentir ou s'interrompre complètement depuis maintenant un an.

d'abord, des conséquences morales pour de nombreux licenciés et bénévoles, lesquels se voient privés de leur activité hebdomadaire, de leur moment de détente et de convivialité qui caractérisent tant nos clubs. Il s'agit, ensuite, des conséquences financières sans commune mesure. Aussi, comme je l'avais dit lors de la première lecture, nous ne pouvons que partager l'esprit et les objectifs de ce texte dans la simplification des relations entre les associations et les collectivités et l'amélioration de leur trésorerie. Toutefois, nous ne pouvons occulter un problème de fond : le recul croissant du financement public des associations. Nous le savons tous sur ces travées, la baisse des ressources des collectivités a entraîné une baisse des financements pour les associations. On le doit d'abord à une baisse significative de la mais aussi à une réforme fiscale venue limiter les marges de manoeuvre de celles-ci. Je ne reviendrai pas sur la réserve parlementaire qu'on a préféré supprimer plutôt que de venir limiter l'usage abusif qui pouvait en être fait par une minorité. conséquent, de plus en plus d'associations se tournent vers le privé. Si nos marges de manoeuvre sur les financements de l'État sont faibles, nous devons accompagner et encadrer ce financement par les acteurs privés. Pour en venir au texte, je rejoins l'avis de la commission : nous devons conserver l'équilibre entre les finances des associations et celles des collectivités. À l'article 1, la suppression de la notion d'excédent raisonnable est une bonne avancée. Son maintien aurait posé quelques difficultés, d'abord dans la définition de ce qu'est un excédent raisonnable, car cela aurait entraîné, en conséquence, une modification des pratiques des collectivités, qui auraient dû faire face à la difficulté de définir avec chacune des associations la hauteur de cet excédent raisonnable.

S'agissant du Fonds de développement de la vie associative, je saluerai, comme lors de la première lecture, l'ouverture de la participation des parlementaires aux collèges départementaux de la commission régionale du FDVA. C'est une décision dont nous devrons nous saisir pour venir appuyer les projets locaux. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le travail mené de concert par les deux chambres aura pris du temps, mais il est à saluer. Il permettra de multiplier les sources de financement des associations, mais également d'accompagner la montée en charge du Fonds de développement de la vie associative que nous appelons de nos voeux. Aussi, les élus du groupe RDSE voteront à l'unanimité ce texte. La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous terminons aujourd'hui l'examen de deux propositions de loi sur la vie associative. Permettez-moi de saluer l'ensemble des acteurs associatifs. Leur engagement nous est précieux, par tous les temps, davantage encore depuis un an. Eux aussi sont en première ligne face à la crise sanitaire et à ses répercussions économiques et sociales ; en première ligne pour lutter contre les inégalités et l'exclusion qui s'accroît ou pour maintenir ou recréer de la solidarité et du lien social, dont nous mesurons particulièrement en ce moment l'importance. Le Sénat avait adopté cette proposition de loi en première lecture le 9 juillet 2019. Notre groupe s'était alors abstenu, le passage du texte en séance en ayant considérablement affaibli la portée. Je tiens donc à saluer le travail de conciliation qui a été fait entre les deux chambres. Voilà des années maintenant que les associations voient leurs financements publics diminuer, alors que, paradoxalement, elles se voient déléguer de plus en plus de missions et de responsabilités. La crise sanitaire a exacerbé cet effet ciseaux et les premières indications sur la baisse inquiétante du nombre d'adhésions dans les associations font craindre une amplification du phénomène. Cette proposition de loi apporte des avancées face à cela. La possibilité de conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée en est une. C'est une suite logique de nos travaux, dès le début de la crise sanitaire, permettant aux collectivités de maintenir leurs subventions, malgré l'annulation d'événements culturels ou associatifs. Saluons, d'ailleurs, l'engagement fort de ces collectivités, aux côtés des associations, dans ce contexte. Concernant l'article 1 , nous sommes satisfaits, madame la rapporteure, que vous ayez obtenu une rédaction de compromis qui permet à la fois de sécuriser les associations et les collectivités en fixant un délai de versement des subventions, et d'introduire la souplesse nécessaire pour que ces collectivités puissent établir des échéanciers de règlement, des conventions. utile tant aux associations pour lancer leurs projets qu'aux collectivités pour les accompagner dans la durée. Cette proposition de loi aura aussi été utile pour faire avancer la possibilité de récupérer les fonds dormant sur des comptes inactifs au bénéfice des associations, même si cela s'effectue par un autre véhicule

satisfait moins de la moitié des demandes de soutien qui lui sont adressées et, je le rappelle, finance moins les réseaux associatifs que ne le faisait la réserve parlementaire, quoi qu'on puisse penser de celle-ci. Nous resterons vigilants à ce que cette bouffée d'oxygène pour les associations ne vienne pas justifier une nouvelle baisse de la contribution de l'État. La rédaction de l'article 5 a été revue par un amendement de notre groupe. En prenant en compte le temps particulièrement long de l'élaboration de ce texte, nous avons cherché à rester dans son esprit initial et à permettre d'évaluer les conséquences,

fragilisé, alors qu'il n'avait vraiment pas besoin de cela. Plus récemment, d'autres mesures sont venues inquiéter le Mouvement associatif, telles que certaines dispositions du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Les associations estiment ainsi que, en s'engageant, lors de toute demande de subvention, à respecter les valeurs et principes de la charte des engagements réciproques, elles prennent une obligation contractuelle suffisamment forte pour qu'il ne soit pas besoin de confirmer cet engagement en signant le contrat d'engagement républicain créé par ce texte. Certaines d'entre elles y voient même une suspicion dangereuse par rapport à leurs activités, alors que, bien évidemment, la très grande majorité des initiatives associatives, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, a précisément pour vocation de consolider

nous voici arrivés au terme d'un processus législatif particulièrement long, qui a permis d'aboutir au meilleur compromis, afin d'adopter la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Les enjeux soulevés par cette proposition sont nombreux et ont nécessité un travail approfondi. Le Sénat partage les préoccupations des auteurs du texte initial, qui actent la baisse continue des financements publics à destination des associations depuis une quinzaine d'années, et souhaitent pallier les difficultés rencontrées par le monde associatif. Rappelons que notre pays compte 1,5 million d'associations et que ce nombre augmente de plus de 2 % par an, selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Les associations sont connues pour les services qu'elles rendent, les causes qu'elles défendent, mais leurs impacts sur le territoire vont bien au-delà. Elles ont un rôle dans le développement des échanges et du lien social. Elles contribuent à l'animation et à l'attractivité du territoire ainsi qu'à l'information, l'éducation et la formation. Ainsi, 76 % des maires considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de coconstruction pour répondre collectivement aux enjeux des territoires. Il y a une forte convergence entre les attentes des maires et les réponses que peuvent y apporter les associations. Ces dernières ont une forte capacité à être à l'écoute de leur territoire et à savoir répondre en cohérence avec les besoins qu'elles y captent. Les associations savent apporter des réponses adaptées aux fragilités prioritaires de leur territoire l'attractivité sur les territoires ruraux et la réduction des inégalités en territoire urbain. La capacité à la fois à réduire les fragilités et à faire émerger de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi adaptés à la spécificité de leur territoire est l'une des grandes valeurs ajoutées des associations. Malgré de faibles moyens, les petites associations, qui représentent 70 % de l'ensemble, jouent un rôle important dans de multiples domaines de la vie sociale. Nous le savons : plus les associations disposent de moyens financiers, plus elles sont en capacité d'agir et de multiplier leurs efforts sur le territoire. Afin de préserver cette richesse, il était nécessaire de garantir les sources de financement, de simplifier les relations avec les autorités administratives et d'accompagner la montée en puissance du Fonds de développement pour la vie associative. Jacqueline Eustache-Brinio, rapporteure de la commission des lois, a été particulièrement attentive à la question de la conciliation des intérêts des associations avec ceux des collectivités territoriales. Le Sénat a voulu, dès la première lecture, enrichir le texte afin de préserver cette relation de confiance. Nous nous félicitons que l'Assemblée nationale ait respecté les modifications apportées par notre chambre, notamment le renforcement des obligations en matière de transparence des comptes, lorsque l'association conserve tout ou partie d'une subvention publique non consommée. Cette disposition assure que les relations conventionnelles avec les collectivités sont équilibrées. par notre collègue Henri Leroy, ont été conservés. Ils permettent aux candidats ayant recours à une association de financement électorale ou à un mandataire physique de reverser l'excédent de leur compte de campagne à des associations d'intérêt général, et non plus seulement à une formation politique ou à une association particulière. Enfin, le Sénat a obtenu la suppression de l'article qui visait à exclure du champ du droit de la préemption les donations de biens immobiliers effectuées au profit des associations et des fondations. Je tiens à saluer l'excellent travail de Jacqueline Eustache-Brinio, qui a réalisé, en parallèle, le rapport sur le projet de loi relatif au respect des principes de la République. Ce dernier établit de nouvelles relations financières entre collectivités et associations, au travers du contrat d'engagement républicain. Je salue également les échanges constructifs qui ont eu lieu avec vous, madame la secrétaire d'État. Les mesures tendant à faciliter la gestion de la trésorerie des associations, telles qu'elles figurent dans la présente proposition de loi, paraissent alors d'autant plus appropriées. Le souci des associations a été entendu. Il a pu être concilié avec l'intérêt des communes, qui doivent pouvoir s'assurer de la transparence financière de l'utilisation des subventions, à l'heure où les budgets sont de plus en plus contraints. Cette proposition de loi arrive à point nommé au moment où, après une année de mise en sommeil en raison de la crise sanitaire et de forte réduction des aides des collectivités, l'activité de nombreuses associations pourra reprendre.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire est parvenue à l'adoption d'un texte commun.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

dans leur diversité. Il est de notre devoir de ne pas laisser les associations seules face à ce risque d'effacement et de délitement de l'engagement des dirigeants et aux conséquences que cela entraînerait, que ce soit sur l'emploi ou sur les solidarités locales. locales. Pour cette raison, le Gouvernement a accompagné les associations tout au long de la crise sanitaire, par des mesures économiques, par leur intégration dans le plan de relance, par des mesures spécifiques aux secteurs les plus touchés et par des mesures sectorielles.

De la même manière, il est absolument essentiel de mettre en oeuvre un cadre bienveillant à leur égard, afin que la responsabilité financière des dirigeants bénévoles susceptible d'être engagée avec de lourdes conséquences personnelles, même en cas de « simple négligence », ne le soit plus. Une fois la crise sanitaire passée, ces mesures devront redonner aux citoyens le goût de s'investir, du monde associatif et des responsabilités associatives, sans qu'ils aient à craindre des conséquences sur leur patrimoine personnel. Cette proposition de loi a également pour ambition de faciliter le renouvellement des dirigeants dont la moyenne d'âge avance. Ce renouvellement ne peut fonctionner que s'il y a transmission et protection. Seule cette garantie permet la pérennité de leurs actions.

Il permettra également de redonner de l'élan, un second souffle à l'engagement des citoyens et des bénévoles, véritable trésor que nous devons protéger, accompagner et reconnaître. Or donner le goût de l'engagement et de la philanthropie commence dès le plus jeune âge et constitue une priorité. Si des initiatives locales existent déjà dans de nombreux territoires, le Gouvernement soutient vivement la sensibilisation à la vie associative dès le collège. J'avais, par ailleurs, déjà soutenu cette proposition proposition dans mon rapport, remis au Premier ministre de l'époque, sur la philanthropie à la française, étant persuadée que celle-ci est nécessaire au développement de l'engagement citoyen. Valoriser le bénévolat et les associations en inscrivant la sensibilisation à la vie associative dans le cadre de l'enseignement moral et civique des élèves de collège et lycée, au même titre que le service civique, est donc plus qu'une nécessité. C'est avec elles que nous construisons un projet de société et que nous dessinons le monde de demain. Poumon de nos territoires, trésor de notre République, les associations font vivre chaque jour des projets et des actions d'intérêt général,

Ce texte est l'illustration parfaite de ce dont notre société a réellement besoin, à savoir un renouveau de l'engagement citoyen, car il représente un espoir pour notre société et notre jeunesse qui doit et peut le porter. En votant ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « plus encore qu'une liberté, l'association est une réalité qui a puissamment contribué à façonner la société française tout au long de ce siècle, à y renforcer la tolérance, la solidarité, l'innovation. Une réalité qui s'affirme [ ...] reflétant, dans toute leur diversité, l'engagement des Français, leur sens de l'action collective, leur souci de solidarité comme d'ailleurs leur volonté d'épanouissement personnel ». Ces mots de Jacques Chirac, prononcés à l'occasion du centenaire de la loi de 1901, sont plus que jamais d'actualité. Je tiens ici à rendre hommage à l'ensemble des bénévoles, des cadres et des dirigeants associatifs, qui, souvent, ne comptent pas leur temps pour faire vivre leurs associations, tisser, maintenir le lien social, animer les territoires. La commission de la culture en a la conviction : la crise de la covid-19 a montré le rôle essentiel joué par les associations. Cependant, la pandémie ne les a pas épargnées : les informations que j'ai pu recueillir à l'occasion de mes auditions témoignent d'une forte incertitude pesant sur le secteur associatif.

En mai et juin 2020, les bénévoles sont revenus, les activités ont repris, l'emploi dans le secteur associatif est reparti à la hausse, alors que le reste du secteur privé continuait à peiner. Mais le deuxième confinement a marqué un nouvel arrêt brutal pour un grand nombre d'associations. Les remontées du terrain témoignent des doutes existants : les conseils d'administration ont du mal à se tenir, il n'est pas sûr que les bénévoles reviennent. La motivation a chuté. En outre, de nombreuses associations employeuses sont menacées de disparition. Or le secteur associatif est un acteur économique important de notre pays : un salarié du secteur privé sur dix y est employé. Ce tableau sombre ne doit toutefois pas masquer certains points de satisfaction et des lueurs d'espoir. Tout d'abord, un fonds d'urgence doté de 30 millions d'euros pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, accessible aux associations, a été instauré par le quatrième collectif budgétaire. Il est opérationnel depuis la fin du J'y vois la reprise d'une recommandation effectuée par la commission de la culture dans ses travaux sur la pandémie de la covid. L'enjeu est désormais de faire connaître ce fonds aux associations concernées. Ensuite, l'élargissement progressif de la vaccination fait émerger de nouvelles questions relatives au mélange de bénévoles et d'un public de vaccinés et de non-vaccinés. Cela témoigne d'une volonté de relance des activités et de la vie associative. Enfin, cette pandémie a montré l'envie de s'engager d'une partie importante de la population, notamment de la jeunesse, ainsi que la nécessité d'accompagner les associations, pour les aider à se développer et répondre aux attentes des nouveaux bénévoles. La proposition de loi en faveur de l'engagement associatif répond à un certain nombre de ces préoccupations et à plusieurs demandes du monde associatif : elle atténue la responsabilité financière des dirigeants des associations en cas de faute de gestion ; elle s'adresse à la jeunesse, afin de mieux lui faire connaître le monde associatif

Lors de mes auditions, il m'a été indiqué que cette mesure représenterait 19 millions d'euros supplémentaires pour 2021. La commission de la culture ne manquera pas de faire un bilan de cette première année d'application, des difficultés rencontrées comme des améliorations possibles. La proposition de loi traduit l'émergence d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans doute ce texte aurait-il pu aller plus loin. La commission a fait le choix d'une adoption rapide pour soutenir un secteur associatif fortement malmené par la pandémie.

Je tiens d'ailleurs à souligner que, si un très large consensus s'est dégagé au sein de notre commission pour une adoption rapide de ce texte, nous sommes également nombreux à noter les bouleversements qui ont ballotté, voire percuté les associations ces dernières années, y compris indépendamment Les associations font partie de notre quotidien et maillent l'ensemble du territoire français. Leur existence, leurs actions semblent aller de soi à chacun. Leurs problèmes et leurs besoins demeurent toutefois trop souvent invisibles. En première lecture, le Sénat avait souhaité faciliter la reconnaissance de leur rôle d'intérêt général au niveau local, mais la disposition proposée posait de nombreuses questions, raison pour laquelle la commission de la culture n'a pas proposé son rétablissement. Toutefois, madame la secrétaire d'État, le monde associatif a besoin de soutien de la part de la Nation. Ces dernières années, le Haut Conseil à la vie associative a fait plusieurs propositions pour améliorer cette reconnaissance. J'espère que vous y serez sensible, tout comme à l'ensemble des interventions des différents groupes politiques sur ce sujet. Le coeur de l'association, c'est l'humain, l'engagement d'un individu en faveur des autres. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. La transmission de la volonté de s'engager d'une génération à l'autre Le texte prévoit une découverte et une sensibilisation dès le plus jeune âge au rôle des associations et au bénévolat. L'encouragement et la reconnaissance du bénévolat étaient également l'objet de plusieurs amendements adoptés par le Sénat en première lecture. Nous n'avons pas souhaité les rétablir en commission, parce qu'ils suscitaient un certain nombre d'interrogations. La situation économique des entreprises a également fortement évolué depuis 2019. En revanche, les représentants d'associations que j'ai pu rencontrer, qu'il s'agisse de têtes de réseau ou d'associations locales, m'ont indiqué la nécessité d'encourager le bénévolat et ont souligné l'investissement en temps des bénévoles. y passent des soirées et, souvent, tous leurs week-ends- je pense aux dirigeants et encadrants des associations sportives, par exemple -ou encore une partie de leurs vacances. D'ailleurs, l'une des inquiétudes des associations porte sur le retour des bénévoles qui auront redécouvert les week-ends et soirées libres de tâches associatives Comme l'a rappelé notre collègue Michel Savin en commission, le statut de bénévole doit être mieux reconnu et valorisé, notamment par des actes. On ne peut en rester là, sans faire de proposition pour l'avenir. Aussi, permettez-moi de conclure mon propos par une proposition, madame la secrétaire d'État : prendre en compte l'engagement associatif dans le calcul de la retraite. Dans notre système de retraite universelle, ce serait une reconnaissance par la Nation d'un don de temps et d'énergie au service de la collectivité fait plus tôt dans sa vie. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le tissu associatif qui maille notre territoire et l'ensemble des associations qui le composent sont au coeur des enjeux pour notre pays. Mobilisant des millions de personnes, les associations font partie du quotidien de nos concitoyens et répondent à leurs besoins sociaux, notamment en entretenant un lien social, d'autant plus important dans les périodes difficiles que nous traversons. Les associations font face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. Le rapport de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif en faisait déjà le constat L'année 2020 a toutefois été particulièrement ardue pour nombre d'entre elles. Le Mouvement associatif a ainsi indiqué que 66 % des associations avaient dû suspendre leurs activités ou revoir leur mode de fonctionnement au printemps 2020 et que près de 30 000 risquaient le dépôt de bilan dès l'automne. Outre l'aspect financier, la crise sanitaire a également touché les associations sur le plan de l'emploi : 55 000 associations indiquaient, en septembre 2020, ne pas pouvoir maintenir leurs effectifs salariés en l'état. N'oublions pas que ces difficultés s'inscrivent dans un contexte déjà en peine, la baisse drastique des contrats aidés- 36 % en 2017 et 50 % en 2018 -ayant fortement affaibli le secteur. La création des associations a connu une baisse de 40 % en 2020 et, dans les secteurs du sport, du loisir et de la culture, les adhésions sont en recul de 25 % à 40 sans parler du bénévolat des seniors, particulièrement vulnérables à la covid-19. Tous ces chiffres représentent autant d'impacts sur le lien social de notre pays. La vie en société place tout être humain, dès sa naissance, dans une relation d'interdépendance avec les autres, et la solidarité constitue, à tous les stades de la socialisation, le socle de la liaison de l'homme aux autres et à la société. Nos associations sont les instruments et les vecteurs de cette socialisation, en particulier de la solidarité nationale. S'associer correspond à s'unir, à faire participer, à former un ensemble, cet ensemble dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. présente proposition de loi ne permet malheureusement que quelques avancées, relatives à l'atténuation de la responsabilité financière des cadres associatifs en cas de faute de gestion à l'éligibilité au service civique des ressortissants algériens ou encore permettant de relever de dix à vingt le plafond de salariés pour pouvoir bénéficier de l'offre de service « impact emploi ». Ces dispositions ont fait l'objet d'un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat dès la première lecture. à l'occasion de la deuxième lecture permet également de voir émerger un consensus concernant les dispositifs de sensibilisation à l'engagement associatif dans le temps scolaire et relatifs aux comptes associatifs en déshérence. À ce propos, je tiens à saluer le travail de mon collègue Jacques-Bernard Magner, qui avait déposé un amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019 tendant à la remise d'un rapport pour étudier les possibilités d'affecter les montants des comptes inactifs des associations au Fonds pour le développement de la vie associative. Cette mesure a depuis été intégrée à la proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations, qui vient d'être examinée par notre assemblée. Quelques réserves peuvent être émises.

Cela soulève également une interrogation quant à la pertinence, pour le Parlement, de légiférer sur le contenu des programmes quand existe un organisme, le Conseil supérieur des programmes, dont la mission principale consiste justement à élaborer les programmes. Une autre réserve concerne la suppression, à l'Assemblée nationale, de la possibilité de dérogation à la limitation du nombre de stagiaires dans les structures associatives. Si cette disposition est protectrice pour l'emploi, en ce qu'elle limite le recours aux stages précaires et mal rémunérés, on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette suppression, notamment dans le contexte de difficultés actuelles du secteur, dont j'ai parlé précédemment, et ce pour une durée limitée, le temps de sortir de la crise sanitaire.

de loi. La parole est à M. Cédric Vial, pour le groupe Les Républicains.

nous devons nous prononcer ce matin sur une proposition de loi en faveur de l'engagement associatif. Quel important sujet ! Nous vivons dans une société qui a une tendance naturelle au repli sur soi et dans laquelle l'individualisme est un comportement de plus en plus partagé. Les interactions avec les autres de nos concitoyens se développent au travers du filtre des écrans et des réseaux dits « sociaux ». Ces relations numériques favorisent bien souvent une forme d'agressivité individuelle et permettent à tout un chacun de se bercer de l'illusion qu'il n'a pas besoin de collectif pour s'exprimer ou pour faire. Nous vivons dans une société où la violence et même l'hyperviolence se développent à une vitesse inimaginable. Cette violence prend de court notre entendement, mais aussi nos autorités, incapables de réactions adaptées. L'issue vers laquelle ce glissement violent de notre société nous entraîne semble tellement irréelle qu'il est plus facile de la nier que d'essayer de l'éviter ou de se préparer à y faire face. Nous vivons dans une société où les inégalités sociales et économiques se creusent. Les divisions entre les gagnants de la mondialisation, de l'ubérisation ou de la nouvelle économie et ceux qui s'en estiment les victimes ou qui en paient réellement les conséquences n'ont jamais été aussi grandes. Nous vivons dans une société dans laquelle de nouvelles fractures territoriales apparaissent : entre le monde urbain et le monde rural, entre les villes et leurs périphéries ... Tout le monde se sent oublié. En réalité, beaucoup vivent leur leur situation comme le résultat d'un mauvais traitement, d'une politique qui sépare les territoires et voudrait leur imposer des modes de vie différents des leurs. Bref, ils se sentent injustement considérés. Nous vivons dans une société qui ne distingue bientôt plus les valeurs des principes, qui ne considère plus l'autorité et n'a que trop peu recours au respect de l'autre, qui pose les croyances individuelles au-dessus des règles de la vie collective. Derrière ce diagnostic, pessimiste- je vous l'accorde, mes chers collègues -et pas assez nuancé- je vous l'accorde également -, il existe tout de même des points positifs auxquels se raccrocher, des comportements à encourager, des valeurs humaines et humanistes, qui laissent à penser que la seule solution n'est pas le déclin si nous savons nous appuyer sur ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Le fait est que l'engagement pour l'intérêt général et l'altruisme sont encore des notions vivantes, qu'il convient de soutenir et de développer. L'avenir de notre monde- ce que certains appellent « le monde d'après » -dépendra pour beaucoup de la générosité dont nous saurons faire preuve dans le monde actuel et face à ses réalités. La vie associative est l'une des principales richesses de notre pays. On estime à 13 millions le nombre de bénévoles présents dans au moins une des quelque 1,3 million d'associations aujourd'hui actives en France. Chaque année, 70 000 associations sont créées, et le nombre de bénévoles était en augmentation ces dernières années. Ces quelques éléments éclairent d'un espoir nouveau le tableau de notre société que j'ai dressé de manière un peu sombre. Pourtant, depuis un an, une partie de ce monde associatif est pratiquement à l'arrêt. La crise sanitaire que nous traversons a révélé à la fois un aspect peu glorieux de notre humanité, mais aussi une capacité à la solidarité, à l'innovation sociale et à la bienveillance sans précédent. Il est de notre devoir d'élus et de citoyens d'encourager ces comportements civiques et solidaires, qui se retrouvent le plus souvent sous la forme d'un engagement associatif. Retrouver, à la prochaine rentrée, un niveau d'engagement bénévole au moins équivalent à ce qu'il était avant la crise, faire retrouver le chemin des clubs aux jeunes licenciés du monde sportif ou culturel : voilà des enjeux majeurs. Il est à notre portée S'appuyer sur les expériences et les nouvelles solidarités qui se sont également exprimées durant cette période, pour construire un monde meilleur et tourné vers les autres, est un autre des enjeux auxquels nous nous devons de répondre. Cette proposition de loi a pour objectif de faciliter et d'encourager l'exercice de fonctions associatives, en atténuant la responsabilité financière des dirigeants associatifs bénévoles en cas de faute de gestion, en sensibilisant les élèves de l'enseignement secondaire à la vie associative ou en relevant de dix à vingt le seuil à partir duquel une association peut bénéficier du dispositif « impact emploi ». Ce programme semble bien maigre par rapport aux enjeux de la vie associative, mais toute mais toute avancée doit être prise en considération. L'engagement désintéressé de millions de bénévoles contribue à donner du sens à notre vie collective. Donner de son temps, de son expérience ou de ses compétences au profit d'une cause, qu'elle soit sociale, caritative, sportive, culturelle ou civique, c'est faire don aux autres d'une partie de soi, et c'est justement cela « faire société ». Il est aisé de réunir un consensus autour de ces valeurs d'engagement,

Nous partageons donc la motivation et les intentions de ce texte, tout en regrettant l'extrême modestie de son contenu. Même s'il est raisonnable de penser que la situation de l'engagement associatif ne sera guère différente après son adoption, l'intention est bonne : toute avancée, aussi minime soit-elle, mérite d'être engrangée tout signe de reconnaissance envers l'engagement associatif, aussi minime soit-il, mérite d'être considéré. C'est si peu, mais c'est déjà quelque chose ! Pour ces raisons, malgré quelques réserves et les regrets que le texte lui a inspirés à l'issue de la première navette parlementaire, notre groupe votera cette proposition de loi.

la crise sanitaire fait vaciller le monde associatif. La plupart des associations culturelles et sportives ont été contraintes de fermer leurs portes et de suspendre leurs activités durant les confinements successifs. Des milliers d'entre elles risquent une cessation d'activité, car leur fonctionnement repose souvent sur l'obtention de subventions, sur la perception de cotisations, sur le bénévolat et sur l'organisation de manifestations. Tout leur modèle économique est mis à mal. La dernière enquête réalisée par Recherches et solidarités indique que la plupart des associations ont dû revoir leur fonctionnement, notamment à travers la mise en place d'outils numériques, pour développer le « télébénévolat Pourtant, la crise sanitaire et l'isolement contraint de beaucoup de nos concitoyens ont démontré la pertinence des actions du secteur associatif pour animer la vie locale et favoriser le lien social. Dans nos villes et nos villages, une association locale est souvent le dernier rempart contre la solitude et la première école de la démocratie. Cette proposition de loi, déposée par Sylvain Waserman, a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

Ce rapport préconisait, entre autres dispositifs, de renforcer l'accès à la formation des dirigeants associatifs et la sensibilisation du public au bénévolat. Plus de quinze ans après sa publication et l'extension du chèque emploi associatif, nous restons dans l'expectative d'une réforme globale du secteur associatif, afin de favoriser son développement au service de la société. Le texte que nous examinons en deuxième lecture contient des mesures visant à encourager la prise de responsabilité associative et l'engagement de la jeunesse. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires soutient cette initiative. Le réseau associatif français compte près de 13 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés, dont l'action est organisée par les dirigeants d'association. Ces derniers manquent trop souvent d'accompagnement technique et de connaissances en matière de gestion comptable et administrative. la proposition de loi, en étendant l'exception de négligence applicable aux dirigeants d'entreprise en cas de faute de gestion conduisant à une insuffisance d'actifs aux dirigeants d'association, permettra de rendre plus attractif l'exercice de responsabilités à titre bénévole.

ainsi que le dispositif tendant à créer un crédit d'impôt pour responsabilité associative. Je regrette que ces dispositions ne soient plus présentes dans le texte que nous examinons, bien que je comprenne les motifs de leur retrait. L'article 2 porte sur la sensibilisation des jeunes au bénévolat, du CM2 au lycée. Je pense que nous devons aller plus loin et étendre les mesures de reconnaissance de l'engagement associatif des étudiants aux lycéens. Enfin, l'article 3 ouvre à bon escient l'accès au service civique aux ressortissants algériens résidant en France. Cette proposition de loi, aux contours modestes, apportera de nouvelles garanties afin de favoriser le renouvellement des dirigeants bénévoles et l'engagement de la jeunesse. Pour aller plus loin, il nous faudrait améliorer la lisibilité fiscale des dispositions applicables aux associations, dont la complexité est souvent un obstacle à leur appropriation. « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière », disait l'abbé Pierre. Le monde associatif est ce sourire adressé à la société, loin de toutes considérations mercantiles, un lieu particulier dans lequel s'exerce la première de nos libertés celle d'agir pour aider son prochain et s'inscrire dans une aventure humaine. À l'heure de la montée des tensions communautaires, l'engagement est un art de vivre. l'« arche d'alliance » décrite par Albert Camus, dont la tâche consiste à éviter que « le monde ne se défasse

Le secteur associatif attend que cette proposition de loi aboutisse rapidement, et, après les mois extrêmement durs que nous venons de traverser, nous espérons son entrée en vigueur le plus tôt possible. En effet, comme la proposition de loi visant à améliorer leur trésorerie, que nous venons de voter, ce texte comporte des avancées très attendues par les associations. d'abord, l'élargissement de l'exception de négligence aux dirigeants associatifs est de nature à rassurer les bénévoles qui s'engagent dans la gestion quotidienne d'une structure. Cela favorisera la prise de responsabilités, parfois lourdes, les fonctions de président ou de trésorier, quand plus de la moitié des associations indiquent qu'elles ont du mal à renouveler leurs instances dirigeantes- vous en avez parlé, madame la secrétaire d'État. l'extension du dispositif « impact emploi » à toutes les associations de moins de vingt salariés, contre dix actuellement, facilitera les démarches administratives en matière sociale et fiscale pour les petites structures. Rappelons que l'ensemble du secteur associatif représente 1,8 million d'emplois en France. Enfin, l'article 1 permettra d'allouer les avoirs des comptes inactifs des associations au FDVA. Ce soutien financier pour accompagner la formation des bénévoles est essentiel.

mis de nombreuses associations culturelles et sportives totalement à l'arrêt. Alors que les contraintes se desserrent tout juste depuis hier, une question se pose : comment faire revenir les adhérents, éloignés depuis parfois un an ? Comment faire revivre les clubs de foot, de chant, de danse ? Ajoutons à cela l'inquiétude au sujet des subventions. Si, en 2020, les collectivités ont été au rendez-vous pour maintenir leur soutien aux associations- il faut le saluer -, les premières remontées pour 2021 sont inquiétantes : les associations craignent parfois de faire office de variable d'ajustement face à la pression qui pèse sur les budgets locaux.

contrat d'engagement républicain obligatoire pour toucher une subvention, contrat d'engagement républicain obligatoire pour recevoir un agrément, contrat d'engagement républicain obligatoire ne serait-ce que pour avoir une salle à disposition Des millions de bénévoles sont désormais suspects. Ce sont 1,3 million d'associations que vous avez regardées globalement comme des niches de l'islamisme radical. Ces associations font pourtant vivre tous les jours la promesse républicaine dans notre pays ! Certaines assurent le travail de lien social dans les quartiers où l'État a fait reculer les services publics. Les mesures proposées dans le texte que nous examinons aujourd'hui sont nécessaires, mais on ne peut pas, d'un côté, louer le rôle primordial et la place des associations dans notre République et, de l'autre, instaurer un carcan qui fait peser une incertitude permanente sur les associations et leurs bénévoles. Le mois dernier, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Mouvement associatif ainsi que des ONG demandaient l'abandon du contrat d'engagement républicain, véritable menace sur la liberté d'association. Aujourd'hui, vous ignorez ces alertes. Mes chers collègues, le monde associatif est un acteur essentiel de notre société, y compris quand, par certaines de leurs méthodes d'engagement, certaines associations nous bousculent, nous alertent, remettent en cause nos certitudes et font avancer la société. Ne les affaiblissons pas. Gardons ce dynamisme associatif qui fait notre grandeur et notre richesse démocratique.

Faciliter l'engagement associatif, tel est l'objet de la présente proposition de loi, examinée elle aussi selon la procédure de législation en commission. Là encore, l'issue devrait être positive. Tant mieux ! mieux ! De quoi parlons-nous ? De l'essentiel. Nous nous adressons, depuis le début de la matinée, à plus de 1,3 million de structures, à un Français sur quatre qui est engagé bénévolement, à près de 2 millions de salariés. Nous parlons de plus de 22 milliards d'actifs et d'un budget annuel de 170 milliards d'euros. Ce tissu associatif remarquable a été soumis, ces derniers mois, à rude épreuve. Il a été en première ligne et mobilisé à chaque instant- je pense aux entités sociales ou sanitaires.

... Finalement, plus d'une association sur deux a perdu des revenus, et probablement des bénévoles, depuis le début de la crise. Deux impératifs s'imposent par conséquent aux responsables politiques que nous sommes répondre présent et simplifier la continuité ou la reprise des activités ; soutenir l'engagement, et ce dès le plus jeune âge. Les députés auteurs du texte- je pense notamment à M. Erwan Balanant, mon collègue finistérien -ont rappelé à juste titre, lors de son dépôt en 2018, que les associations répondent pleinement « aux besoins sociaux et sociétaux » et participent au maintien des liens entre les personnes. Je le disais, nous parlons de l'essentiel. Cette proposition de loi, comme la précédente, fait écho à plusieurs objectifs défendus dans un rapport remis par le Mouvement associatif au Premier ministre,

Il est temps que nous ayons en France une politique publique digne de ce nom, ambitieuse et moderne, pour soutenir la création, la vitalité et la croissance de la vie associative. » Il ajoutait : « Il y a un enjeu crucial à retrouver de la cohésion sociale, d'une part, et à investir dans les transitions vers une économie plus juste et plus soutenable, d'autre part. ajouter à cela la fragilisation occasionnée par la crise sanitaire. C'est pourquoi nous saluons la position de la commission de permettre une adoption rapide du texte pour soutenir le monde associatif fortement malmené. fortement malmené. En première lecture, la Haute Assemblée a intégré plusieurs dispositions qui ont été votées conformes par l'Assemblée nationale ou qui ont fait l'objet de simples modifications rédactionnelles. Ce dispositif vise, finalement, un seul objectif : encourager la prise de responsabilité associative et tenir compte de la réalité du monde associatif et de ses fortes contraintes. de loi ont également souhaité valoriser le bénévolat en inscrivant la sensibilisation à la vie associative dans le cadre de l'enseignement moral et civique des élèves du secondaire, au même titre que le service civique. Madame la secrétaire d'État, ces mesures viennent en complément du texte discuté à l'instant, que vous aviez déposé, en tant que députée, à la suite des annonces faites à destination du monde associatif. Favoriser le bénévolat, l'engagement, c'est préserver la richesse du tissu associatif français. C'est aussi maintenir ou créer des activités, des services de la vie dans nos territoires ruraux. Je veux

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à quelques jours des cent vingt ans de la fameuse loi fondatrice du droit à la liberté d'association, c'est un honneur pour un radical de porter la voix du groupe du RDSE. Cette loi consacre encore aujourd'hui le tissu associatif français, animé par plus de 13 millions de bénévoles. C'est une richesse exceptionnelle, qui a encore prouvé sa force, sa vitalité et son utilité au cours de la crise sanitaire et économique que nous traversons. Le monde associatif est au coeur du quotidien de nos concitoyens, qu'ils soient bénévoles ou bénéficiaires. Il a démontré son rôle d'amortisseur social. Nous savons tous ici combien ces 1,3 million de structures contribuent à l'équilibre de nos territoires, en oeuvrant largement à leur attractivité.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 Pourtant, les associations ont souffert de la réduction du nombre d'emplois aidés, de la diminution des dotations aux collectivités ou encore de plusieurs réformes fiscales, qui ont affecté le niveau des dons. La conjoncture difficile dans laquelle évolue aujourd'hui le monde associatif doit retenir toute notre attention. Cela apparaît même crucial au regard de son utilité sociale et économique. Les pouvoirs publics doivent donc agir de façon à valoriser et à encourager le dévouement d'une grande partie de la société civile. Le Gouvernement et les collectivités territoriales l'ont bien compris cette année en apportant le soutien nécessaire à la survie d'un grand nombre d'associations. Il faut aussi souligner la générosité accrue de nos concitoyens. La portée de cette proposition de loi est certes modeste, mais elle apporte une aide non négligeable à l'essor de la vie associative. Parmi les obstacles rencontrés figure notamment la trop lourde responsabilité financière des dirigeants des associations en cas de faute de gestion. Les auteurs de ce texte y ont répondu à l'article 1. Cette insécurité juridique est source de préoccupations dans le milieu associatif et freine le renouvellement des instances dirigeantes. Je ne parle pas de la nécessaire vigilance à apporter aux activités lucratives qui, sous couvert d'associations de circonstances, ne rémunèrent que le seul promoteur ou les proches du responsable d'association. L'article 2 permet la mise en place d'un module théorique et d'un support méthodologique destinés à aider les enseignants dans la présentation de la vie associative. Il est crucial de mieux sensibiliser les élèves de collège et de lycée dans le cadre de l'enseignement moral et civique et, ainsi, de les inciter à s'engager afin de former le vivier du milieu associatif et de citoyens de demain. C'est l'occasion également de relever l'esprit de coopération qui a animé nos deux assemblées parlementaires pour la construction de ce texte. Ainsi, le Sénat a relevé à vingt le nombre de salariés permettant à une association de bénéficier de l'offre de service « impact emploi » de l'Urssaf, qui assouplit les formalités de gestion salariale. Cette disposition, reprise à l'Assemblée nationale, va dans le bon sens en faveur d'un accompagnement plus fort de la part de l'administration. Pour toutes ces raisons, nous nous associons pleinement aux propositions contenues dans ce texte. Cependant, il faut aller au-delà, car, sans le soutien de l'État et des collectivités territoriales, le secteur non lucratif, auquel sont confiées de plus en plus de missions de service public, ne peut agir de manière efficace. Pour donner un nouveau souffle au bénévolat et au tissu associatif, peut-être serait-il temps de mieux les accompagner en supprimant les trop nombreux formulaires bureaucratiques et en valorisant davantage le service civique Ce texte nous permet d'envoyer un signal fort aux associations et de reconnaître qu'elles constituent un vecteur essentiel de l'engagement citoyen et un moyen d'action à la portée de tous au sein de la société civile. Et puis, n'oublions pas que la vie associative permet aussi aux retraités de continuer à être des citoyens « actifs ». Leur disponibilité et leurs compétences sont une richesse.

C'est proprement ne valoir rien que de n'être utile à personne », disait Descartes. L'engagement associatif en est une belle

dont nous débattons aujourd'hui. Ce texte permettra notamment d'atténuer la responsabilité financière des dirigeants associatifs en cas de faute de gestion en leur étendant l'exception de négligence. Ce

en cas de condamnation, des conditions matérielles de soutien administratif constituent de véritables avancées. Souhaitons que cette protection permette à davantage de bénévoles de prendre des responsabilités, car, chacun le sait, il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui acceptent de siéger au bureau des associations ou de les présider. L'élargissement des conditions pour prétendre au dispositif « impact emploi » de l'Urssaf est aussi une avancée. Établir les formalités administratives d'embauche ou des fiches de salaire demande des compétences particulières. Même si l'on peut saluer la montée en compétence des militants associatifs, leur offrir de tels services nous semble tout à fait utile. Je salue également l'ouverture du service civique aux jeunes ressortissants algériens. Ce dispositif fait partie de ceux qui peuvent participer à la construction de la citoyenneté. Chacun voit bien également l'intérêt de donner aux jeunes une meilleure connaissance du rôle des associations et du tissu associatif local afin de les éveiller à l'engagement

Cette rémunération permettrait sans doute à davantage de salariés de devenir responsables associatifs. On le sait bien, prendre la direction d'une association implique différentes missions- rencontres, échanges, actes de gestion -qui ont souvent lieu lors des horaires de travail. Ce n'est pas sans raison que nombre de nos associations sont dirigées et animées par des retraités. Ils y ont évidemment toute leur place, mais favoriser l'implication des actifs amènerait, là encore, neuf. Le congé associatif existe bien, mais il est aujourd'hui synonyme de perte de revenu pour des salariés, ce qui en limite l'utilisation par la plupart des responsables associatifs. Cette proposition de loi ne suffira malheureusement pas à résoudre la crise de l'engagement, qu'on ne peut mettre sur le seul compte du développement de l'individualisme et du repli sur soi que les confinements successifs auront sans doute amplifié. La précarisation croissante, le développement de formes brèves de travail, la multiplication des horaires décalés, les temps de transports allongés laissent peu de place à l'engagement citoyen, quel qu'il soit. Si vous me permettez une petite digression, je dirai que le peu de considération à l'égard des corps intermédiaires, un mode de gouvernance de plus en plus solitaire au plus haut niveau du pouvoir, le dos tourné aux propositions citoyennes pourtant sollicitées, les entorses de plus en plus fréquentes à nos libertés fondamentales fondamentales ne contribuent pas à donner goût à l'engagement- au contraire ! Eh oui ! Pourtant, dans ce contexte peu réjouissant, la crise semble avoir accéléré l'engagement des jeunes, avec un fort besoin de se sentir utile et, quelque part, de trouver sa place dans la société. Maintenant, il faut transformer La crise sanitaire a aussi accentué la crise des associations : alors que, depuis vingt ans, 70 000 associations étaient créées en moyenne chaque année, on annonce une baisse de 40 % en 2020. Les adhésions

tout en continuant à travailler, avec tous ceux qui le souhaitent- je sais qu'ils sont nombreux ici -, sur le statut de bénévole, qui doit être mieux reconnu et valorisé, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes. La parole

remercie également notre rapporteur, Pierre-Antoine Levi, de son excellent travail. Pour la commission d'enquête de l'Assemblée nationale chargée, en 2014, d'étudier les difficultés du monde associatif, le renouvellement des dirigeants bénévoles est la première difficulté recensée par les associations : 53 % d'entre elles indiquent avoir du mal à renouveler leurs instances dirigeantes. Rappelons que les ressorts principaux de l'engagement sont avant tout la volonté d'être utile à autrui et à la société, de lutter contre les injustices. Les valeurs essentielles en sont la fraternité et la solidarité. Mais les bénévoles d'aujourd'hui, sur qui repose largement le fonctionnement des associations, souhaitent aussi que leur engagement leur apporte un épanouissement personnel et qu'il donne un sens à leur vie. vie. Pour ces raisons, le mode de fonctionnement des associations et l'appétence à s'engager se devaient d'être interrogés. En ce qu'elles jouent un large rôle de vecteurs de lien social, synonymes de cohésion territoriale et sociétale, il était important que les associations, qui pallient aussi parfois les manquements de l'État en jouant un rôle de service public, et le monde associatif en général soient l'objet du texte qui nous préoccupe aujourd'hui afin de corriger ce biais carentiel d'engagement.

L'un des maillons essentiels en est d'ailleurs le dirigeant bénévole, qui, outre un engagement sans faille en termes de disponibilité, doit notamment disposer de compétences solides en matière fiscale et juridique, eu égard aux responsabilités dont il est débiteur. Il était donc primordial de lutter contre une insécurité juridique délétère et de lui offrir un cadre stable en atténuant sa responsabilité financière en cas de faute de gestion due à de simples négligences. Je salue l'abondement du FDVA, qui va dans le bon sens. Je rappelle que le Haut Conseil à la vie associative estime à 100 millions d'euros les sommes qui pourraient ainsi ainsi être mobilisées. Par ailleurs, et de manière plus large, cette proposition de loi vise à favoriser l'engagement associatif auprès des plus jeunes en permettant la mise en place d'un module théorique et d'un support méthodologique pour aider les enseignants dans la présentation de la vie associative et aider ainsi les élèves de collège et de lycée à s'engager et à développer une fibre d'engagement citoyen. c'est bien d'éveil dont il est question : il faut que nos jeunes aient une réelle connaissance et soient largement sensibilisés à ce type d'organisation, en leur permettant de s'engager pour une cause et de et de faire vivre une passion. Malgré les engagements positifs de cette proposition de loi, la fatalité de l'existant est réelle et de nombreux points restent en suspens et doivent nous interroger en termes de viabilité, d'efficacité et de pérennisation de la vie associative. Le secteur associatif a été rudement éprouvé par les mesures prises depuis le début du quinquennat avec le retrait des contrats aidés, la diminution des moyens publics, l'impact sur la générosité de la suppression de l'ISF

associées à une valorisation timorée de l'engagement associatif. Tous ces aspects continueront de peser négativement sur l'engagement associatif et de grever les actions mêmes des associations. Or il faut justement répondre aux besoins spécifiques de toutes les associations : celles qui emploient plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de salariés, mais aussi les plus petites, qui jouent souvent un rôle décisif dans la vie économique et sociale au niveau local.

en direction du milieu associatif. Il est d'une impérieuse nécessité de développer une reconnaissance de l'engagement associatif au-delà de ce qu'il est aujourd'hui possible de faire et qui, je le précise, est très largement méconnu.

et la reconnaissance du caractère d'intérêt général des associations par le préfet. Malgré cela, et dans un souci de pérenniser rapidement les avancées qu'offre cette proposition de loi, le groupe Union Centriste, au nom duquel j'interviens aujourd'hui, votera ce texte. Je mets aux voix,